Monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est avec émotion et tristesse que nous avons appris, dans la soirée d'hier, la disparition du Président Valéry Giscard d'Estaing. Au nom du Sénat tout entier, je souhaite rendre hommage, dans notre hémicycle, à un homme d'État au parcours exceptionnel, qui a profondément transformé notre pays. Valéry Giscard d'Estaing a occupé successivement les plus hautes fonctions de la République, chaque fois de manière précoce.

et il le reste jusqu'en 1966. Il occupe de nouveau ce poste de 1969 à 1974, sous le mandat du Président Georges Pompidou, avant d'être élu à la présidence de la République. Valéry Giscard d'Estaing incarne alors l'avenir, le changement. Il admire profondément le général de Gaulle, même s'il lui arrive d'avoir avec celui-ci des désaccords politiques, qui ont commencé par le « oui,

Candidat à l'élection présidentielle, il affronte les électeurs avec une image- celle de la modernité -, un projet- la société libérale avancée -, un slogan- « le changement sans risque » -et quelques belles formules, comme : « Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Président de la République, à 48 ans, il entreprend une vaste politique de réformes. Il souhaite aller vers une démocratie renforcée plus de libéralisme, et faire entrer de plain-pied notre pays dans ce qu'il qualifie de « monde moderne ». D'abord, pour signifier, de manière symbolique, un changement de style, l'injure au chef de l'État cesse d'être un délit. Puis vient l'élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel, changement capital, dont même Michel Debré admet, dans ses, le caractère positif

à 18 ans ; la loi qui humanise le divorce, au travers de la notion de consentement mutuel ; la généralisation de la sécurité sociale à tous les Français ; la réforme de l'ORTF

mais également avec la loi sur l'interruption volontaire de grossesse- un moment très important -, défendue avec tant de noblesse et de courage par Simone Veil ; il manifeste ainsi sa résolution et son esprit d'indépendance.

poste de président du Parlement européen, à Strasbourg, lui doit beaucoup et concrétisera l'influence et l'action de la France. Le rôle décisif qu'il joue dans la construction européenne lui vaudra d'être, plus tard, désigné président de la Convention qui proposera une Constitution pour l'Europe. Après son échec de mai 1981, il éprouve un sentiment d'injustice qu'il décrit dans son livre. Il revient alors au sein de son Auvergne, où il gravit à nouveau les échelons de la vie politique, la députation et la présidence du conseil régional. La pensée de Valéry Giscard d'Estaing, telle qu'elle s'exprime dans, est une exhortation à l'apaisement politique, un appel à substituer le dialogue au conflit, la négociation à la lutte ; une inspiration qui vise à conjurer la fatalité de la seule bipolarisation. Valéry Giscard d'Estaing était attaché au bicamérisme il demeure le seul Président de la République à être intervenu au sein même de cet hémicycle ; c'était le 27 mai 1975, pour le centenaire du Sénat de la République. À cette occasion, évoquant la III République, Plus circonspect que la Chambre [des députés], moins sensible qu'elle à la séduction d'idéologies non encore éprouvées au contact des réalités, le Sénat a apporté dans la gestion des affaires publiques le concours de l'expérience et de la sagesse » ; comme un écho au discours de Bayeux, prononcé, en 1946, par le général de Gaulle. Nous garderons tous le souvenir de sa grande intelligence, d'un Président moderne et réformateur, d'un militant de la construction européenne.

afin que nous soyons, non pas « deux Français sur trois » mais trois Français sur trois à croire en la République et en ses valeurs, dans la diversité que nous formons. En ce jour où la Haute Assemblée va examiner les crédits de la mission « Outre-mer », je ne peux m'empêcher d'évoquer également l'intérêt que Valéry Giscard d'Estaing portait aux outre-mer. Il fut ainsi le premier Président de la République à se rendre dans l'île de Wallis

ont trouvé un écho singulier dans les différents territoires d'outre-mer, notamment pour les femmes et pour la jeunesse. Le surnom de « prince qui a fendu les océans

Dans l'océan Atlantique, il a marqué les Antilles, dans un moment compliqué socialement ; on se souvient d'un déplacement tendu mais au cours duquel il a su trouver les mots pour renouer avec la population et lancer des initiatives diplomatiques importantes. Cela a ainsi permis de positionner la Martinique et la Guadeloupe au coeur de grands sommets internationaux, notamment pendant la guerre froide,

mais aussi pour l'énergie nucléaire ainsi que pour la place de la France en Europe. Cette érudition, cette capacité à penser vite, cette curiosité, cette bienveillance, quoiqu'un peu taquine, je dois bien l'avouer, nous ne les oublierons pas. C'est vrai, le Président Giscard d'Estaing a occupé différentes fonctions. Il aimait à me dire qu'il avait eu beaucoup de plaisir à exercer des fonctions exécutives locales,

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2021, adopté par l'Assemblée nationale (projet

je veux tout d'abord rappeler la vocation particulière de la mission « Outre-mer » : favoriser le rattrapage, par les territoires ultramarins, de leur retard économique et social par rapport à l'Hexagone. Cet objectif se manifeste notamment par le fait que plus de 90 % des crédits demandés pour 2020 étaient des dépenses d'intervention. Le rattrapage de cet écart persistant constitue le défi majeur de la mission.

la comparaison avec les données de la France entière montre également une meilleure résistance des économies ultramarines, en raison principalement du poids plus important, dans ces territoires, du secteur non marchand. La crise économique constitue néanmoins un facteur supplémentaire de ralentissement de la convergence des économies ultramarines avec l'Hexagone, l'un des principaux objectifs, je le

Le principal point de vigilance sur lequel je souhaite attirer votre attention est la sous-exécution importante dont cette mission fait l'objet. Il s'agit d'une question centrale et récurrente, souvent mise en avant par les gouvernements successifs pour expliquer la situation des outre-mer ces derniers seraient presque responsables de leur situation parce que les crédits existent mais ne seraient pas consommés faute d'ingénierie locale.

La sous-consommation s'explique également par la situation financière de nombreuses collectivités locales, qui ne disposent pas de l'épargne nécessaire et qui souffrent d'un déficit du compte de fonctionnement. Il est crucial de les remettre à flot financièrement, afin qu'elles puissent s'inscrire dans le plan de relance. Concernant le logement, la question du manque d'ingénierie ne devrait pas se poser, dans la mesure où les opérateurs immobiliers ont de très bons services en la matière. En outre, la disponibilité du foncier fait souvent défaut avant de prévoir des crédits destinés à la construction, il conviendrait d'en prévoir pour l'aménagement du foncier. Dans certains territoires, en effet, le foncier est rare et cher. Dans d'autres, comme en Guyane, le foncier existe, mais il doit être aménagé et il serait judicieux d'avoir des crédits pour cela, à l'image du fonds régional d'aménagement foncier et urbain. Action Logement m'a également fait part d'une sous-consommation des crédits, pourtant disponibles. Cette sous-consommation des crédits budgétaires est d'autant plus préoccupante que, en 2019, le Gouvernement avait demandé la suppression de 170 millions d'euros de dépenses fiscales en outre-mer : suppression de la TVA non perçue récupérable (TVA NPR) et recentrage de la réduction d'impôt sur le revenu dans les territoires d'outre-mer. Il s'était toutefois engagé à utiliser les gains budgétaires dégagés pour abonder le fonds exceptionnel d'investissement (FEI) et financer les dépenses visant à favoriser le développement économique des territoires. J'avais appelé l'attention du Sénat, à l'époque, sur le fait que les dépenses budgétaires, contrairement aux dépenses fiscales, n'offrent aucune garantie dans la durée et peuvent faire l'objet de sous-consommation.

Le programme 138, « Emploi outre-mer », rassemble les crédits visant à compenser, auprès des organismes de sécurité sociale, les exonérations spécifiques de cotisations patronales. En 2019, le dispositif d'allégements et d'exonérations de charges patronales de sécurité sociale spécifiques aux outre-mer a été modifié, afin de répondre entièrement aux dispositions de l'article 86 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, qui actait la suppression du crédit Cette réforme avait entraîné, en 2019, une augmentation de plus de 42 % des crédits affectés à la compensation de ces exonérations de charges. Ces derniers connaissent, en 2021, une hausse de 6,4 % par rapport à ceux qui Nous tenons à rester vigilants quant à la fiabilité de ces prévisions, parce que la baisse de l'activité qui résulte de l'épidémie et le recours important au chômage partiel sont susceptibles d'entraîner une sous-exécution importante. En pareil cas, il nous paraît important que les crédits restants soient affectés à d'autres dépenses de la mission. Sur le fond, je tiens à le dire, les nouveaux paramètres du régime issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 n'ont pas pleinement compensé les effets de la suppression du CICE à 9 %. Cela a entraîné une augmentation du coût du travail en Guyane, alors même que ce territoire subit une forte concurrence extérieure et reste particulièrement vulnérable par rapport à l'économie informelle. Les conséquences économiques de l'épidémie devraient être de nature à susciter une réflexion sur un éventuel élargissement du barème de compétitivité renforcée à de nouveaux secteurs, afin d'apporter un soutien suffisant aux territoires ultramarins. ailleurs, le projet de loi de finances pour 2021 ne comprend aucune évolution en matière fiscale concernant les outre-mer, alors que ce levier aurait été pertinent pour mobiliser l'épargne face à la crise.

Comme chaque année, je rappelle que la mission ne concerne qu'une part faible de l'effort de l'État en faveur des outre-mer. C'est particulièrement vrai aujourd'hui, puisque les territoires ultramarins devraient bénéficier d'au moins 1,5 milliard d'euros dans la cadre du plan de relance national. Une vigilance particulière s'imposera néanmoins quant à la déclinaison territoriale de ce plan et à la bonne exécution des crédits. En outre, dans la mesure où une partie importante des dépenses dépend d'appels à projets, aucune garantie ne peut être apportée à ce stade quant au montant dont les outre-mer bénéficieront réellement.

les chiffres sont têtus ! Malgré la crise, l'effort de l'État en faveur des outre-mer est réel. Il est en hausse non seulement sur cette mission, mais aussi, de manière transversale, sur l'ensemble des missions du projet

En cette période extraordinaire, au sens premier du terme, plutôt que de joutes verbales décapantes, il nous faut relever le défi de l'efficacité et de l'efficience des moyens déployés par l'État et par chacune de nos collectivités, pour apaiser l'urgence sanitaire et conjurer le mauvais sort économique, que la division de nos énergies risque d'aggraver.

trouver des solutions pour gérer les urgences. Comme dans l'Hexagone nos populations vivent dans l'espoir d'une année 2021 à l'aune d'un ou plusieurs vaccins salvateurs, mais aussi et surtout d'un rebond économique impératif, urgent et crucial. Nous avons Nous avons été beaucoup plus exposés qu'ailleurs à l'arrêt brutal du tourisme et des transports, qui a produit des effets directs et indirects dévastateurs sur des marchés étroits et concentrés. Le seul secteur du tourisme a chuté jusqu'à 90 % dans certaines collectivités ultramarines. L'urgence est à la reconsolidation de nos économies, à la formation des hommes pour les préparer à cette reprise indispensable et à la stabilité des dotations publiques alimentant nos moteurs économiques éparpillés sur tous les océans du monde.

Ce programme rassemble, en plus des crédits destinés aux exonérations de charges sociales, les crédits du service militaire adapté (SMA), qui constitue une formidable opportunité, une deuxième chance offerte par la République à nos jeunes en difficulté d'insertion. Ses crédits sont en augmentation de 4 % en AE et il fait l'objet d'un ambitieux plan dit « SMA 2025 », qui prend pleinement sens en ces temps de redressement face à la crise.

tous les observateurs l'attestent : la mission « Outre-mer » doit quitter le podium de la sous-exécution ou sous-consommation- cela est fonction des hémisphères d'analyse. Je sais que d'autres voix s'exprimeront différemment, mais l'ajustement du niveau des CP relève, selon moi, de la mécanique financière logique et implacable : il est fonction des décaissements escomptés sur l'année concernée, pour faire simple, comme pour toutes les lignes s'exécutant de manière pluriannuelle. Nous avons pour défi un regain d'engagements, de nouvelles contractualisations, de nouvelles concrétisations réelles, effectives et à un rythme plus élevé de portée contracyclique. Que faire ? Si l'accusé se nomme ingénierie, redoublons d'appui aux collectivités territoriales, notamment en matière de gestion de projets. Des efforts ont été faits sur ce plan. Néanmoins, ne détournons pas le regard. La simplification des procédures et des normes, l'accessibilité des informations ainsi que la territorialisation des budgets forment autant de gages de souplesse ou d'agilité, pour employer une formule du moment, comme le relève la Cour des comptes.

Le FEI maintient son fort niveau de dotation à 110 millions d'euros, pour accompagner l'équipement de nos territoires. En 2021, l'effort sera maintenu en AE pour les contrats de convergence et de transformation, le futur contrat de développement et de transformation en Polynésie française en cours de finalisation et le contrat de développement en Nouvelle-Calédonie.

Des retards de paiement ont aussi été relevés. La parole de l'État doit pourtant reposer sur un socle de confiance inébranlable. Nous relevons que le montant cumulé des charges à payer relatives à ces contrats s'élevait, en fin de gestion 2019, à 3,6 millions d'euros, ce qui constitue le plus bas niveau historique et traduit la volonté de ce gouvernement d'honorer les engagements de l'État, quel que soit celui qui les a pris par le passé. Programmons ce que nous pouvons payer et engageons ce que nous pouvons réaliser : voici le maître-mot de nos prochains contrats, selon les principes de différenciation mais aussi de responsabilité commune dans un respect mutuel.

est vrai qu'ils sont à un niveau très inférieur à celui qui a été constaté jusqu'en 2017 et qu'ils sont frappés d'une sous-exécution chronique, comme cela a été souligné. Les crédits prévus et dépensés en 2021 devraient donc se trouver largement inférieurs aux besoins, alors que le rythme souhaité de construction de logements sociaux est estimé à plus de 15 000 par an relative à l'égalité réelle outre-mer. Voilà un fait tout aussi têtu qu'incontestable. Le sénateur que je suis ne saurait affirmer d'autre axe que celui de la différenciation en associant les énergies locales,

Je tiens à le remercier pour son engagement et son dévouement à nos océans de France. Chers collègues, avec quelques points d'attention, mais aussi avec responsabilité, je constate que nos budgets de la mission « Outre-mer » sont en augmentation, malgré certaines sous-exécutions chroniques. Notre défi, au-delà de la course aux crédits, est de remporter la bataille de l'efficacité pour gagner au champ de la responsabilité. C'est dans un partenariat franc et constructif avec l'État, qui est à nos côtés en ces temps de crise comme lors de la relance prochaine, que nous réussirons tous. Je me joins donc à l'avis de mon collègue Georges Patient en invitant le Sénat à adopter ces crédits et l'État à les exécuter avec nos collectivités.

Monsieur le président, monsieur le ministre,

À cet égard, monsieur le ministre, pouvez-vous confirmer l'engagement pris en 2019 de recycler, chaque année, les prélèvements supplémentaires provoqués par la suppression de dispositifs fiscaux qui bénéficiaient aux ménages et aux entreprises ?

C'est bien cette volonté que le Sénat a exprimée en adoptant un amendement tendant à prévoir 2,5 milliards d'euros, apportant du reste un démenti au préjugé d'outre-mer budgétivores, d'autant que les crédits affichés restent, trop souvent non consommés. face au risque d'effondrement du secteur marchand, de flécher ces crédits du plan de relance territoire par territoire. Nous vous alertons sur les risques du « premier arrivé, premier servi ». Un grand nombre de très petites entreprises ayant des projets utiles et créatifs ne sont pas outillées pour déposer rapidement des dossiers. Sur certains territoires, un tiers des TPE ignorait purement et simplement les dispositifs du premier confinement. C'est dire combien la gestion et la numérisation doivent être soutenues. Je termine par un impératif : saisir la chance historique qui se présente pour le logement ultramarin. En effet, les financements de relance mobilisables vont bien au-delà des crédits budgétaires ; avec les plans d'investissement volontaire d'Action Logement et de CDC Habitat, on est sans doute proche des sommes investies par l'État pendant quinze c'est-à-dire plus de 3 milliards d'euros. Le véritable défi est d'activer ces fonds en redynamisant un secteur qui a un puissant effet d'entraînement sur les économies de nos outre-mer. L'objectif doit être de développer sur place des filières intégrées : aménagement, nouveaux matériaux, construction, habitat et traitement de l'amiante. Selon nous, ce mouvement doit être impulsé par des mécanismes et des opérateurs qui doivent adopter le modèle de l'entreprise formatrice. face à des taux de chômage vertigineux, il faut intégrer la jeunesse ultramarine, qui regorge de jeunes talents. Monsieur le ministre, l'acte de construire et ses ramifications ont également besoin d'un encadrement mieux adapté. la Cour des comptes vient de souligner l'existence d'exigences normatives « sans réel rapport avec les réalités locales », faisant ainsi écho aux préconisations de notre délégation sénatoriale Tout aussi réaliste, le haut-commissaire au Plan déplore que l'État, avec les règles actuelles, entrave même ses propres actions. Le moment est venu de sortir de ce carcan.

comprennent qu'un peu plus d'un dixième de l'ensemble de l'effort budgétaire de l'État à destination des territoires ultramarins. La commission des affaires sociales est à la fois satisfaite du maintien du niveau des crédits de la mission, au-dessus du seuil symbolique de 2,5 milliards

de Martinique, de Guyane, de La Réunion ainsi que de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Monsieur le ministre, notre commission s'est émue de ce que les exonérations Lodéom, principal outil du budget dont vous êtes l'ordonnateur, semblent non pas faire l'objet d'une stratégie d'ensemble, mais plutôt revêtir la forme d'un secours en urgence porté, à différents secteurs. J'en veux pour preuves l'heureuse intégration de la production audiovisuelle dans le régime de compétitivité renforcée à la suite de la fermeture de France Ô

Le programme « Conditions de vie outre-mer » comprend, d'une part, le financement budgétaire et fiscal de la politique de logement, et, d'autre part, diverses actions budgétaires aux vocations disparates, qui ont toutes pour point commun de prévoir d'importants transferts aux collectivités territoriales. Dans

dans un rapport récent la pertinence discutable d'un financement reposant de plus en plus sur la dépense fiscale, là où l'intervention budgétaire serait sans doute plus pertinente. Elle les difficultés issues de l'intervention, sans ordre de bataille, de dix-neuf organismes de logement social (OLS) pour l'ensemble des territoires ultramarins.

». En effet, il s'agit d'augmenter uniquement les crédits de ceux qui ont été précédemment dans l'incapacité de les dépenser, au détriment de ceux qui en ont trouvé par eux-mêmes le bon emploi. Sous ces réserves, et en renouvelant son souhait que les crédits sociaux de la mission « Outre-mer » fassent l'objet d'un pilotage plus fin et plus adéquat, la commission des affaires sociales a donné un avis favorable à leur adoption.

Les crédits de paiement pour 2021 sont ajustés à ce qui devrait être effectivement dépensé. En outre, 70 % des crédits de la mission devant être disponibles dès janvier,

la construction et la rénovation des infrastructures ; le soutien à l'emploi et à la formation ; l'accompagnement des collectivités territoriales. Les crédits alloués à la mission augmentent ainsi nettement par rapport à 2020 : une hausse de 6,39 % en autorisations d'engagement et de 2,64 % en crédits de paiement. En matière de construction et de rénovation des infrastructures, 2021 constituera la deuxième année de mise en oeuvre du plan Logement outre-mer 2019-2022. Un effort important sera fait en matière de construction d'écoles. D'autres dispositifs sont également maintenus, comme l'aide aux ménages de Guadeloupe et de Martinique pour l'acquisition de terrains dans la zone des cinquante pas géométriques ou la suite de l'opération de rénovation du quai de croisière de Saint-Pierre-et-Miquelon. En matière de soutien à l'emploi et à la formation, 84 % des crédits du programme « Emploi outre-mer » sont, cette année encore, destinés à compenser les exonérations de charges patronales accordées aux entreprises ultramarines. Ce dispositif a été étendu en 2019 à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Dans les collectivités du Pacifique, des mesures d'insertion professionnelle spécifiques sont mises en place, notamment pour les chantiers de développement local en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Quant au service militaire adapté, il a montré toute sa pertinence lors de la crise sanitaire. Une nouvelle compagnie vient d'être créée à Bourail en Nouvelle-Calédonie, tandis que des opérations de rénovation structurante auront lieu à La Réunion et en Polynésie française.

Des plateformes d'aide à l'ingénierie à destination des collectivités ont ainsi vu le jour à Mayotte et en Guyane en 2020, mais il existe également des dotations spécifiques, notamment en Polynésie française, pour renforcer les moyens d'intervention des territoires. Pour terminer, je souhaite rappeler que les crédits portés par la mission « Outre-mer ne constituent qu'environ un dixième de l'effort total de l'État en faveur des territoires ultramarins, qui se monte à 24,47 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 24,13 milliards d'euros en crédits de paiement. L'ensemble de ces éléments a conduit la commission des lois à émettre un avis favorable à l'adoption de ces crédits.

qu'ils ne représentent qu'une minorité des engagements de l'État dans nos territoires. Pour rattraper notre retard structurel sur l'Hexagone, dans presque tous les domaines, il est nécessaire que le « réflexe outre-mer » que nous réclamons régulièrement ici devienne la règle, et ce dans tous les ministères. Il s'agit là d'une demande, non pas de rattachement de crédits liés à l'agriculture ou à la culture à la mission « Outre-mer », mais bien de mise en place d'une collaboration efficace entre tous les services du Gouvernement. Le but étant le déblocage des fonds nécessaires pour l'alignement équitable de nos territoires sur l'existant hexagonal. de prendre l'exemple des fonds CIOM, qui, malgré une promesse claire du Président de la République, ont pris plus d'un an pour être augmenté, à la suite d'un imbroglio autour de la provenance des fonds entre votre ministère et ceux de l'agriculture et du travail. Il n'est pas normal que des annonces faites lors de l'examen des missions du PLF restent aussi floues pendant si longtemps. J'en tiens pour responsable la mauvaise coordination des différents ministères sur des questions pourtant essentielles pour nous. Tout cela concernant non pas directement la mission « Outre-mer », mais bien le fonctionnement général des politiques publiques dans nos territoires, je vais tout de même parler rapidement du détail de ce budget. L'accent mis, cette année, sur le logement social constitue, bien évidemment, une bonne chose, puisque nombre de nos concitoyens vivant dans des conditions extrêmement précaires, rendues parfois plus difficiles par un accès à l'eau aléatoire et des infrastructures insalubres.

Concernant les aides aux entreprises et à l'emploi, le dispositif d'exonération des charges patronales atteint, aujourd'hui, son rythme de croisière, bien que l'année écoulée ne constitue pas le meilleur indicateur de son efficacité. À cet égard, il est aussi nécessaire

entre les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, entre la théorie de la politique publique et sa transcription sur nos territoires bien particuliers. J'illustrerai là aussi mon propos par un exemple passé. Le FEI, Le FEI, annoncé il y a deux ans comme une solution exceptionnelle dans les stratégies de développement de nos territoires, justifiant par ailleurs la fin de l'exonération de la TVA NPR, finance aujourd'hui bien peu de projets d'envergure, en tout cas pas à la mesure de l'ambition affichée au départ. Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, comme nombre de mes collègues, je suis satisfait de l'augmentation du budget de cette mission. Ce sentiment est toutefois édulcoré par un peu de frustration et de doute. Au-delà de cette ambitieuse budgétaire de 6 %, nous avons besoin d'une refonte globale de nos plans d'investissement pour notre santé, notre culture et notre production agricole. Or, cette ambition, nous ne la voyons toujours pas arriver. Nous avons tout de même de bonnes raisons de vous faire confiance

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette discussion budgétaire s'inscrit dans un contexte particulier, car la crise sanitaire liée au covid-19 frappe douloureusement nos territoires d'outre-mer. Les inquiétudes de nos concitoyens ultramarins sont très importantes et l'évolution de la situation constitue une préoccupation de chaque instant. Comme vous le savez, les territoires ultramarins sont déjà fragilisés par une balance commerciale déficitaire, des taux de chômage deux à trois fois plus élevés qu'en métropole, une insularité et un éloignement géographique favorisant la vie chère. Aussi, dans ce contexte inédit de pandémie, les crédits de la mission « Outre-mer » doivent être, plus que jamais, mobilisés au service de nos territoires ultramarins. C'est donc avec satisfaction que je constate une légère augmentation par rapport à l'année 2020. Ces crédits s'élèvent ainsi, pour 2021, à 2,68 milliards d'euros en autorisations d'engagement et à 2,34 milliards d'euros en crédits de paiement,

À cet égard, je regrette que l'action de l'État à destination des territoires ultramarins manque quelque peu d'ambition en s'inscrivant dans la continuité des années précédentes.

de la ligne budgétaire qui lui est consacrée, la portant à 224 millions d'euros en autorisations d'engagement. Il s'agit d'un signal positif envoyé aux territoires ultramarins en matière de lutte contre l'habitat indigne et d'accès au logement. Cela permettra de poursuivre la mise en oeuvre du plan Logement outre-mer et d'accompagner les stratégies territoriales des établissements publics fonciers et d'aménagement de Guyane et de Mayotte. En deuxième lieu, je tiens à évoquer les difficultés du secteur touristique, qui représente, en moyenne, plus de 18 % du PIB- emplois directs et indirects. À l'heure de la deuxième vague pandémique, les faibles chances de reprise du secteur semblent définitivement compromises.

Par conséquent, la relance pérenne de l'économie ultramarine doit reposer sur une meilleure adaptation des dispositifs d'urgence à ces territoires. et dernier lieu, je souhaite mettre l'accent sur la nécessité d'améliorer l'emploi et la compétitivité des entreprises ultramarines- elles sont, à 95 % des TPE et des PME -, notamment grâce à l'allégement des cotisations patronales. Les moyens budgétaires prévus pour ce dispositif, en hausse de 6,6 % par rapport à 2020, représentent 1,5 milliard d'euros. Je salue ce levier important qui vient soutenir les nombreuses petites entreprises ultramarines, moins résistantes à un choc économique d'une telle ampleur et d'une telle durée. À titre d'exemple, sur l'île de la Réunion, les entreprises ont considérablement réduit leurs embauches et 4 300 emplois ont été détruits depuis le début de la crise sanitaire. Monsieur le ministre, mes chers collègues, bien qu'il manque, une fois de plus, d'ambition,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la mission budgétaire « Outre-mer » s'articule autour de plusieurs axes : le soutien à l'emploi, l'insertion socioprofessionnelle des jeunes, les actions de formation en mobilité, le logement social, l'effort d'équipement des territoires et l'éducation et l'accompagnement des collectivités territoriales. Néanmoins, beaucoup des crédits utiles à l'outre-mer proviennent d'autres ministères. Au regard des besoins, cette architecture budgétaire morcelée est dommageable. Les territoires ultramarins accusent des retards sur les plans économique et social. À titre d'exemple, le PIB par habitant est près d'une fois et demie supérieur dans l'Hexagone qu'en Guyane. Il y est près de trois fois plus élevé qu'à Mayotte. Les effets de la crise économique et sociale, résultat de la pandémie de covid-19 en outre-mer- je pense notamment à l'effondrement du tourisme -, viennent s'ajouter à une situation déjà très précaire.

le premier poste budgétaire de celle-ci est l'action Soutien aux entreprises, qui vise à financer les dispositifs d'allégements et d'exonérations de charges patronales de sécurité sociale spécifiques aux outre-mer.

La baisse d'activité liée au covid-19 provoque un recours massif au chômage partiel. Ce dispositif réglant déjà la question des charges patronales de sécurité sociale, il est probable que les crédits ou du moins leur hausse soient surévalués. Alors qu'ils auraient pu être fort utiles ailleurs, ces crédits risquent d'être utilisés pour éponger la dette de la sécurité sociale. La sous-exécution des crédits est un problème récurrent de la mission budgétaire « Outre-mer », comme plusieurs de mes collègues l'ont rappelé. La ligne budgétaire unique, qui finance le logement en outre-mer, en est le témoin. Son taux d'exécution s'est élevé à 90 % en autorisations d'engagement et 78 % en crédits de paiement. Pourtant, les besoins sont réels ! Le ministère des outre-mer évaluait le nombre de ménages ultramarins en attente d'un logement social à 60 000 en 2019. Dans un rapport de septembre dernier, la Cour des comptes évoquait « 80 % d'ayants droit pour 15 % de bénéficiaires ». Dans son analyse, elle explique que la diminution des autorisations d'engagement dans la ligne budgétaire unique aura un impact négatif dans le futur sur le total des prêts accordés et sur le nombre de logements sociaux produits. Cependant, il nous est proposé une ligne budgétaire unique aux autorisations d'engagement réduites de 2,7 %. Pour résumer la situation, des crédits alloués au logement ne sont pas consommés pendant que la demande de logement social augmente ! Pis, le budget qui nous est proposé va contribuer à cette La question du logement n'est pas le seul rendez-vous manqué par le Gouvernement. La liste en est longue : maigre pouvoir d'achat, précarité, faiblesse de la politique de l'eau et de la politique de mobilité, absence d'une politique de retour sur le territoire. Par ailleurs, le Gouvernement ne tire pas ne tire pas les conclusions des années précédentes. Le service militaire adapté, le SMA, par exemple, a montré toute sa pertinence dans l'intégration des jeunes sur le marché du travail. Pourquoi ne pas lui allouer davantage de crédits ?

Monsieur le ministre, j'ai sans doute mal regardé, mais je ne parviens pas à évaluer, ni dans les crédits de la mission « Écologie » ni dans les crédits spécifiques du plan de relance, la part des fonds pour la biodiversité qui est fléchée vers l'outre-mer. Pourriez-vous m'éclairer à ce sujet ? De manière générale, ne serait-il pas préférable que la protection de la biodiversité ultramarine fasse l'objet d'un programme spécifique de la mission budgétaire « Outre-mer » ? Cela nous semblerait plus transparent et plus efficace pour bénéficier de fonds pérennes.

Toutes les formations de cet hémicycle ont pris la mesure de l'urgence de la situation et vous rendent service. Utilisez ce levier pour lever le gage et, ainsi, doubler les crédits de votre ministère Dans l'attente de votre réussite, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s'abstiendra sur les crédits de la mission. La

J'insisterai plutôt sur la mise en place du plan de relance, dont 1,5 milliard d'euros sont dédiés aux outre-mer, avec des interrogations légitimes sur leur déclinaison par territoire. Je reviendrai également sur le programme 123, relatif aux « Conditions de vie outre-mer », sans omettre évidemment l'impact de la crise sanitaire dans nos territoires. Enfin, je prendrai brièvement mon archipel pour exemple, afin de rappeler que, si nous voulons relancer une dynamique dans l'outre-mer, il est essentiel que l'État fasse confiance aux élus locaux, qui disposent d'une légitimité démocratique. Quel que soit le budget examiné, cette crise sanitaire n'aura laissé personne indemne. C'est tout particulièrement vrai de nos territoires ultramarins, déjà fragilisés par de nombreux déséquilibres structurels.

Plus encore que les collectivités de l'Hexagone, qui connaissent évidemment elles aussi leurs propres difficultés, les collectivités ultramarines, en moins bonne santé financière avant l'épidémie de covid-19, subissent de plein fouet une double crise sanitaire et économique qui affecte leurs budgets locaux, même si je note que des mesures de compensation sont prévues dans le plan de relance, Concernant les « Conditions de vie outre-mer », j'ai tout d'abord une pensée particulière pour nos collègues de Mayotte et la Guyane, qui ont été durement frappées durant la crise. Sur le volet économique, je vous renvoie aux propositions contenues dans le rapport intitulé « Urgence économique outre-mer à à la suite de la crise du covid-19 », où nous appelions, au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer, à un meilleur accompagnement des collectivités dans la crise. Il s'agirait de favoriser une relance territorialisée, avec une adaptation des dispositifs nationaux aux réalités de notre tissu entrepreneurial, afin de construire, pour l'avenir, un modèle de développement plus résilient.

collègues, de faire un parallèle avec les syndromes post-traumatiques liés aux événements climatiques. La délégation sénatoriale aux outre-mer a formulé des propositions tendant à la mise en place de dispositifs de prise en charge psychologique.

En ce qui concerne le plan de relance, nous veillerons bien évidemment avec intérêt à sa déclinaison territoriale. Au-delà des montants alloués, je rejoins tous mes collègues, qui indiquent que l'ingénierie et le pilotage seront déterminants pour une réussite collective. Tous les observateurs sont d'accord pour dire que, si nous voulons que la relance soit pérenne et efficace, elle doit s'appuyer sur une réelle adaptation des dispositifs à nos territoires, au titre de la différenciation territoriale.

Nous subissons une situation de blocage institutionnel anormale, contre laquelle je ne peux que me dresser. Jamais je n'aurais cru devoir le faire à cette tribune et à ce moment précis, mais c'est ainsi. Quand on prétend rechercher des partenaires de confiance, il faut être loyal et ne pas saborder à dessein des projets majeurs de développement du territoire. Bien sûr, ce que je dénonce se fait de manière très intelligente, sous couvert d'un État républicain, mais la population n'est pas dupe.

L'écrivain Jérôme Leroy a déclaré : « En politique avoir raison n'est rien, convaincre est tout. » Comme de nombreux compatriotes, je ne suis pas du tout convaincu de certains choix de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon, monsieur le ministre. Au-delà de ces considérations strictement locales, je vous indique que le groupe RDSE votera les crédits de la mission « Outre-mer

pour créer un nouveau programme, intitulé « Plan pour l'égalité réelle outre-mer » et doté de 2,5 milliards d'euros. C'est à peu près le montant des crédits de la mission « Outre-mer » que nous examinons aujourd'hui. L'objectif de cette mission est de réduire les écarts entre l'Hexagone et les collectivités d'outre-mer. C'est ambitieux, mais impératif. Lorsque l'on parle d'égalité républicaine, nous avons l'ambition que les valeurs qui s'y rattachent soient partagées sur tout le territoire français, peu importe la distance qui sépare Paris de Papeete, Cayenne ou Pointe-à-Pitre. Les crédits de la présente mission sont insuffisants pour répondre à cet enjeu de l'égalité républicaine. Certains soulignent l'évolution de l'enveloppe globale. Certes ! Pour notre part, nous souhaitons insister sur la baisse des crédits de paiement de l'action Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle, sur la diminution de 5 % de ceux du programme « Conditions de vie outre-mer », de quasiment 3 % de l'action Logement ou encore de 10 % de l'action Aménagement du territoire. Nous parlons de crédits de paiement. nous souhaitons alerter, comme malheureusement chaque année, sur la sous-consommation des crédits de la mission « Outre-mer ». Cette non-utilisation de crédits ne justifie en rien la réduction des moyens alloués. Les difficultés à engager les dépenses de cette mission sont inacceptables. Nous demandons au Gouvernement d'agir à ce sujet. Le Parlement ne peut voter des crédits qui ensuite ne sont pas

Cette sous-exécution chronique concerne notamment le logement, dont les crédits sont très inférieurs au niveau constaté jusqu'en 2017 et bien en deçà des besoins ressentis en outre-mer. Il y a 69 432 demandeurs de logements sociaux et les besoins de logements sociaux sont évalués à plus de 10 000 par an. La crise du logement en outre-mer est nourrie par la forte pression démographique, la rareté du foncier, l'urbanisation rapide, la pauvreté des ménages et l'insalubrité. Pourtant, la commission des finances dénonce un niveau de crédits « historiquement bas La crise touche de manière différenciée nos collectivités d'outre-mer, mais elle aggrave les inégalités. Rappelons que la part des jeunes de 18 ans en difficulté de lecture varie entre 30 % et 75 % dans les départements d'outre-mer, contre 10 dans l'Hexagone. Le taux de chômage est deux à trois fois plus élevé qu'en métropole. Les personnes les moins qualifiées y sont surexposées. Par conséquent, la formation des jeunes doit être améliorée, et il faut renforcer les moyens de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, d'autant plus que ses dispositifs sont déstabilisés par la crise. Les effets de la pandémie creusent les écarts

coûtent en moyenne 12 % plus cher en outre-mer, et même jusqu'à 28 % à La Réunion, où un quart des habitants vivent avec moins de 867 euros par mois. La pauvreté s'ajoute à cette « vie chère ». Le taux de pauvreté atteint ainsi 77 % à Mayotte, contre 14 % en France métropolitaine, où seul le taux de pauvreté de la Seine-Saint-Denis est à peu près comparable à celui de certains territoires ultramarins. L'épidémie implique d'appliquer des règles sanitaires de base, comme se laver les mains. comment en faire un geste naturel lorsque l'on n'a pas d'eau au robinet ? Une réelle politique de l'eau doit être mise en oeuvre en outre-mer, où la vétusté des réseaux entraîne, au quotidien, des coupures et des contaminations. Monsieur le ministre, des crédits nous sont présentés, mais leur lecture ne nous inspire aucun enthousiasme. Nous savons bien que nous abordons un sujet transversal, touchant l'ensemble des ministères, mais votre rôle est essentiel pour faire entendre la voix de l'outre-mer auprès du Gouvernement. Les enjeux sont de taille

Aussi, chaque année, le Sénat salue l'effort financier global de l'État en faveur des outre-mer sur l'ensemble des programmes. La mission « Outre-mer » définit trois priorités principales, afin de contribuer à la reprise économique qui suivra la crise sanitaire. Cette crise a largement affecté l'économie de nos îles, sur des secteurs aussi importants que le BTP, le tourisme ou encore le commerce. Elle a également touché les publics vulnérables que sont les personnes âgées, les porteurs de handicap, les familles. Je veux aussi insister sur les conséquences de cette période difficile

outre-mer. La politique du logement social en outre-mer est bipède : elle est constituée, d'une part, par les aides directes- les aides à la pierre -, et, d'autre part, par les aides à la personne. L'équilibre du secteur ne peut tenir qu'en renforçant ces deux composantes.

Aussi, au-delà de l'attention que vous portez aux aides directes, monsieur le ministre, nous vous demandons de ne pas fragiliser les ménages, leur solvabilité et, par ricochet, les opérateurs et entreprises qui construisent nos territoires. Vous engagez-vous à nous garantir que, en dehors de la base des ressources prévue par la réforme, les critères d'octroi des aides au logement à caractère familial et social ne seront pas revus outre-mer ? Notre regret à tous vient bien de la sous-consommation des crédits LBU, comme le soulignaient les rapporteurs spéciaux de la commission des finances. Il conviendrait de s'interroger sur ce point avec précision, car il n'est pas normal que de telles sommes soient sous-consommées, alors que nos populations sont dans le besoin.

simplifier et rendre ces fonds accessibles aux TPE et PME, dont de récentes études ont souligné la faiblesse en matière de compétences et d'organisation administrative.

ministre, que vous allez vous impliquer dans ces dossiers. Bien évidemment, le groupe UC votera les crédits de la mission outre-mer.

C'est l'occasion d'insister sur les actions prioritaires à retenir pour nos territoires, afin de réduire le retard persistant avec l'Hexagone. Le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités, publié le 26 novembre dernier, vient nous le rappeler avec force

Cette année, l'examen de la mission présente un caractère particulier du fait de la crise de la covid. L'éloignement, l'insularité, la petitesse des marchés font que les outre-mer sont frappés de plein fouet et voient leur économie vaciller. Aucun secteur n'est épargné : BTP, tourisme, restauration, services, événementiel ... Pour la seule île de La Réunion, ce sont 4 300 emplois qui ont été détruits depuis le début de la crise, malgré les aides diverses mises en place par l'État. Le milliard et demi d'euros du plan de relance consacré en 2021 et 2022 aux outre-mer est le bienvenu. Cependant, comme le rappelle fort justement la commission des lois dans son rapport pour avis, il conviendra « d'être vigilants quant à la consommation concrète de ces crédits, puisqu'une partie d'entre eux dépendra d'appels à projets et rien ne peut garantir dès à présent que ces crédits seront effectivement consommés dans nos territoires ultramarins J'en arrive à l'examen des crédits de la mission pour 2021, qui s'établissent à 2,68 milliards d'euros en autorisations d'engagement et à 2,44 milliards d'euros en crédits de paiement. Les crédits 2021 du programme 138, « Emploi outre-mer », augmentent de 107 millions en AE et 94 millions en CP. Les crédits du programme 123, « Conditions de vie eux une hausse de 55 millions en AE et baissent de 31 millions en CP. Monsieur le ministre, je tenais à saluer certaines annonces et certaines avancées effectuées lors de l'examen des crédits alloués à l'outre-mer à l'Assemblée nationale. Je pense, tout d'abord, à l'augmentation de 3 millions de 3 millions d'euros des dispositifs en faveur de la continuité territoriale, permettant notamment un abondement et une modification des critères d'éligibilité de la « continuité funéraire », ainsi qu'un élargissement du dispositif à la fin de vie. ensuite à la hausse de 8,7 % de la LBU, qui passe à 224 millions en AE, mais aussi à la mise en place de nouveaux contrats avec les collectivités territoriales en difficulté et, enfin, au passage de l'audiovisuel en secteur de compétitivité renforcée.

Monsieur le ministre, je veux étayer mon propos en revenant sur un sujet auquel je tiens et qui est relatif à la continuité territoriale. J'avais déposé un amendement, hélas déclaré irrecevable au titre de l'article 40 à ce que l'aide destinée à financer une partie des dépenses afférentes au transport aérien de corps puisse bénéficier aux familles qui ont perdu un enfant étudiant ou stagiaire à l'étranger, car de nombreux cursus universitaires rendent ces expériences internationales obligatoires.

je souhaite insister sur trois points importants pour l'île de La Réunion. En premier lieu, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d'affaires du secteur a chuté de 40 % en dix ans et a atteint, en 2019, son niveau le plus bas depuis plus de vingt ans. Il est regrettable que l'Assemblée nationale ait supprimé, en nouvelle lecture du PLFSS, la disposition votée par le Sénat permettant aux entreprises du BTP de bénéficier du régime de compétitivité renforcée de manière temporaire. Cette mesure aurait permis au secteur de faire face et de tenir jusqu'à la relance de l'activité, qui est prévue pour la mi-2021. En deuxième lieu, je souhaite insister sur la nécessité d'anticiper l'évolution démographique de nos populations liée au vieillissement. Ainsi, si l'une des trois priorités de la mission « Outre-mer » pour 2021 est la construction et la rénovation des infrastructures, ne faudrait-il pas réfléchir à un fléchage d'une d'une partie des crédits LBU vers la construction de résidences pour personnes âgées à taille humaine, en développant un mode d'habitat innovant adapté à nos modes de vie

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'interviens aujourd'hui pour la première fois en discussion générale dans cet hémicycle, en tant que sénatrice nouvellement élue. C'est une grande émotion, d'autant qu'il s'agit de l'examen de la mission « Outre-mer » du projet de loi de finances. C'est aussi votre premier passage budgétaire en tant que ministre des outre-mer, cher Sébastien Lecornu. Cela renforce mon émotion, car je connais votre sensibilité ultramarine. Je ne reviendrai pas sur l'examen d'ensemble de la mission, qui a déjà été largement évoqué par nos rapporteurs, que je remercie. certains points qui me tiennent à coeur. La Guyane est un territoire frappé de nombreux handicaps structurels, au premier rang desquels son étendue géographique, qui induit l'éloignement et l'isolement de bon nombre de ses habitants. La population guyanaise est jeune, frappée par un taux de chômage élevé et une insuffisance de formation et de qualification professionnelle. J'apprécie donc l'effort porté sur le service militaire adapté, qui est une grande réussite. En Guyane, la création de la troisième compagnie de formation professionnelle et la construction d'un plateau pédagogique constituent une excellente nouvelle. Concernant le programme 123, un effort budgétaire sans précédent est porté sur l'éducation. Je m'en félicite. Le plan d'urgence Guyane et des dotations spécifiques sont importants. permettez-moi d'émettre le souhait que, l'an prochain, à l'instar de ce qui est prévu cette année pour Mayotte, la Guyane puisse bénéficier de nouvelles constructions scolaires, car nos structures sont actuellement insuffisantes et ne permettent pas l'accueil de tous les enfants. Le logement social fait également l'objet d'un effort important, au travers de la LBU. C'est une nécessité absolue, tant cette question est cruciale, en particulier pour la Guyane. La mise en oeuvre de l'opération d'intérêt national en Guyane répond à un impératif. Nous attendons beaucoup de ce dispositif. De même, le renforcement de l'accompagnement de l'État, nécessaire pour la réalisation des plans de développement stratégique de l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane, se traduit par une augmentation bienvenue de l'enveloppe du un grand merci, monsieur le ministre, pour l'aide accrue de l'État en matière de logement et d'aménagement du territoire en Guyane. La croissance démographique dans l'ouest guyanais impose des orientations nouvelles dans tous les domaines, par exemple en matière de santé. Nous aurons notamment besoin de votre appui auprès du ministre de la santé pour la création, unanimement souhaitée, d'un service de réanimation au centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Je reviendrai vers vous sur ce sujet. Pour finir, je dirai un mot sur la question économique. Le soutien au microcrédit en Guyane est précieux.

Je vous remercie de nouveau, monsieur le ministre. Et bien évidemment, notre groupe votera ce budget. La Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les années se suivent et se ressemblent, hélas ! Un hémicycle quasi désert, des lignes budgétaires déjà arrêtées et convenues et des élus qui vont s'acharner des heures entières à tenter de faire comprendre l'évidence et à réclamer le meilleur pour leurs pays. Ils seront tous là, tous présents, bravant kilomètres et risques sanitaires, rappelés à l'ordre par ce sens évident du devoir qui les anime.

Serais-je donc gagnée par la résignation ? Oui, peut-être. Par une forme de résignation qui remporterait la partie contre la détermination et l'optimisme ? Il y a certainement un peu de cela

Tous les jours, il faudra donc se battre aux côtés de nos compatriotes frappés par des indicateurs désastreux. Je me contenterais d'un seul, qui est éloquent : 30 % de la population martiniquaise vit au-dessous du seuil de pauvreté, soit un Martiniquais sur trois C'est pour ces personnes que je continue de venir ici. C'est pour elles aussi que je tente inlassablement de réclamer le meilleur. Et ma demande n'est pas une demande pour plus d'argent, plus de subventions ou plus de moyens financiers. Je viens vous demander, monsieur le ministre, de faire preuve d'ambition. Je viens vous demander une lucidité pour trouver les voies d'un vrai changement de l'approche de nos pays dits « d'outre-mer ». Je sais que vous le pouvez. Chaque année, au dernier trimestre, nous vivons des moments totalement anxiogènes. Que nous réservera cet exercice budgétaire ? Que va-t-on encore changer, faire évoluer, faire disparaître ? Chaque exercice budgétaire est une course à l'information, aux auditions, à l'effarement aussi provoqué par telle ou telle mesure. Et souvent on en sort sonnés, sonnés par les vraies injustices, qui font hurler de douleur des pans entiers

et, record d'incompréhension battu, la suppression de la défiscalisation sur la réhabilitation sociale des logements. J'en oubliais presque la taxe sur le rhum, censée punir les vilains alcooliques que nous serions ! Cette instabilité qui nous épuise, cette instabilité ne rassure pas, cette instabilité qui rajoute de la difficulté à la difficulté.

avec le temps. Il faut de la visibilité pour l'initiative entrepreneuriale : il faut de la visibilité pour les collectivités. Dans ces marchés très contraints, chaque décision a des répercussions, des effets domino qui créent souvent des désastres. Nos entrepreneurs sont épuisés d'être chahutés en permanence. Ouvrez le champ des possibles ! Nous avons les idées, nous savons ce qu'il faut faire. Une fois de plus, les années se suivent et se ressemblent. Nous aurons droit à ces démarches traditionnelles, à nos déclarations et à nos inlassables amendements dont on connaît le sort d'avance- « défavorable

Nos pays sont marqués du sceau de l'inactivité- vous connaissez les chiffres -et j'ai pris l'habitude de dire ici, sans être un grand Grec de l'économie, que l'inactivité coûte forcément plus cher que la mise en activité. Comment pouvons-nous renverser la table, changer de paradigme, voir les choses autrement ? Osons parler port franc, osons parler zone franche globale, osons reparler d'une défiscalisation ambitieuse. Je ne saurais terminer sans vous appeler personnellement à prendre à bras-le-corps le sujet de l'hôpital et de l'accès aux soins à la Martinique. Les conditions d'accueil et l'accès à la santé sont indignes : on meurt à la Martinique, faute de soins, de médecins. L'hôpital de Trinité est une ruine insalubre. insalubre. Il y a des décisions à prendre, et vite, pour doter le nord de la Martinique, le tiers du pays en termes de population, d'un outil qui soit digne de la République. Plus largement, un plan santé est nécessaire.

ce budget n'appellera pas d'observation particulière de ma part. En effet, vous le savez, la collectivité ne bénéficie pas de dotations de l'État. Elle lui verse, en revanche, 2,6 millions d'euros par an au titre de la Cette dernière, du reste, a fait l'objet d'un effacement pour l'année 2018 après le passage de l'ouragan Irma. La collectivité en sait naturellement gré à l'État. Les entreprises de l'île bénéficient, quant à elles, des exonérations de patronales dont les crédits sont inscrits à la mission « Outre-mer » que nous examinons aujourd'hui. Le dispositif applicable à Saint-Barthélemy tient compte de la structure particulière de notre économie, quasi monosectorielle, et de son environnement concurrentiel.

À cet égard, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour vous alerter sur la situation du, seule publication hebdomadaire et gratuite de l'île, car les critères du décret d'aide exceptionnelle à la presse du 13 novembre dernier l'excluent du bénéfice de cette mesure. Or, à terme, sous les effets cumulés de la crise sanitaire et de la réforme des annonces légales, ce journal pourrait purement disparaître. Aussi, monsieur le ministre, je vous serais reconnaissante si une attention particulière pouvait être accordée à cette situation. En dehors de ces aspects budgétaires, qui méritaient, me semble-t-il, d'être évoqués, cette discussion est surtout l'occasion de m'adresser à vous, monsieur le ministre, au titre de la vocation interministérielle de vos fonctions, pour vous demander de relayer les préoccupations de la collectivité, essentiellement relatives à l'aménagement de la décentralisation et à la mise en oeuvre de son projet différencié. La première de ces préoccupations concerne le domaine de la sécurité sociale et des établissements médicaux de l'île. Comme vous le savez, depuis 2017, les missions relevant de la sécurité sociale ont été confiées à la Mutualité sociale agricole, la MSA, qui les assure par le biais de la caisse de prévoyance sociale, la CPS, de Saint-Barthélemy. il n'avait pas été jugé opportun de mettre en place un conseil d'administration ni de doter la caisse de la personnalité juridique. Toutefois, son fonctionnement largement satisfaisant depuis sa mise en place effective en 2017 et son élargissement au régime social conduisent aujourd'hui à souhaiter la redéfinition de son organisation, afin d'y associer plus étroitement et formellement la collectivité. Cela se justifie non seulement par ses compétences- fiscalité, logement, action sociale -, mais aussi par son implication financière dans le fonctionnement des structures de santé de l'île. Le président Bruno Magras avait d'ailleurs eu à alerter le Gouvernement sur la situation déficitaire de l'hôpital et de l'Ehpad, en dépit du concours de la collectivité. S'il en était besoin, la crise sanitaire a mis en lumière cet engagement,

en matière de sécurité sociale et de santé. L'étroitesse du territoire et sa dépendance à l'extérieur à de nombreux égards commandent de faire des choix pertinents en ce qui concerne les politiques publiques mises en oeuvre. Si la compétence en matière de sécurité sociale est une priorité, il n'en que la collectivité souhaiterait, à terme, se rapprocher du régime d'autonomie qui soit le plus abouti possible, tirant les leçons de la pratique du statut actuel. Elle appelle donc de ses voeux une révision ambitieuse des dispositions constitutionnelles, laquelle ne saurait être menée qu'en solidarité et en concertation avec les autres collectivités ultramarines. Je garde espoir que nous puissions aboutir à une position commune, qui, je l'espère également, trouvera en vous un relais, voire un défenseur, au sein du Gouvernement.

Au titre de la rénovation des réseaux d'eau et d'assainissement et de la production d'eau potable, on atteint 50 millions d'euros en crédits de paiement sur deux ans, soit 15 millions d'euros pour l'année 2021.

Le renforcement de la compétitivité des entreprises, notamment dans leur environnement régional, se décline avec une baisse des impôts de production, avec l'amélioration du capital des TPE-PME et avec le soutien à la filière tourisme-appel à projets d'innovation. De plus, je tiens à relever l'adoption, par l'Assemblée nationale, de deux amendements significatifs pour nos territoires. Le premier vise la création de contrats d'accompagnement pour les communes en difficulté dont les efforts de redressement L'objectif de ces contrats est de résoudre l'écart structurel entre recettes et dépenses, comme l'avait préconisé le rapport de décembre 2019 du sénateur Georges Patient et du député Jean-René Cazeneuve sur les finances des communes, des départements et des régions d'outre-mer.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la mission que nous examinons ce matin se voit dotée de crédits en nette augmentation, une hausse de 13,6 % par rapport à 2020, pour s'établir à 2,68 milliards d'euros en autorisations d'engagement et à 2,34 milliards d'euros en crédits de paiement. face à une baisse d'activité de l'ordre de 30 % dans l'ensemble des outre-mer pendant le premier confinement, l'ampleur de la crise dépendra de la rapidité de la reprise. Dès lors, je salue le milliard et demi d'euros du plan de relance national en direction des outre-mer.

Je tenais ce matin à attirer l'attention sur les indispensables aides à la mobilité dédiées à la continuité territoriale, afin que la crise sanitaire ne soit pas synonyme d'enclavement territorial et d'assignation à résidence. nous le savons bien, les outre-mer dépendent des échanges extérieurs, notamment les liaisons aériennes- les premières à avoir subi la crise sanitaire et économique, avec 60 % de trafic en moins entre mars 2019 et mars 2020. Certes, le recours au télétravail, l'enseignement à distance et l'e-santé démontrent l'importance du numérique pour assurer la résilience des territoires. C'est un point important. D'ailleurs, les nouveaux moyens dédiés aux investissements du plan France Très haut Débit ne devront pas oublier les outre-mer, mais contribuer à accroître leur couverture numérique. Toutefois, le besoin de formation, l'importance du tourisme et les questions d'approvisionnement imposent d'assurer cette continuité territoriale. l'accompagnement des collectivités territoriales dans la conduite de leurs projets des plateformes d'aide à l'ingénierie, dont une première évaluation démontre l'efficacité. Ce soutien aux collectivités ultramarines sera indispensable pour les appels à projet du plan de relance.

que l'eau est indispensable pour les gestes barrières et constitue un enjeu d'autonomie- autonomie sanitaire, dans un premier temps, un renforcement des capacités médicales, et autonomie alimentaire, dans un second temps, défi qui pourra être relevé en aidant les agriculteurs et pêcheurs affectés par la crise.

c'est avec une certaine émotion que je m'exprime pour la première fois à cette tribune où d'importantes personnalités ont pris la parole pour la défense des valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité. En cette période où l'extrémisme, l'intolérance et le racisme doivent être combattus au quotidien avec fermeté, je sais que, ici, quelles que soient les travées où nous siégeons, nous lutterons pour le maintien de ces valeurs et leur transmission aux générations futures. Nous abordons aujourd'hui l'examen des crédits de la mission « Outre-mer ». Je ne reviendrai pas sur le détail des chiffres, différents orateurs l'ayant fait avant moi. À l'heure où notre pays tout entier est frappé par une crise sans précédent,

Nous le savons tous, les effets de la crise sanitaire liée à la covid-19 ont eu un effet dévastateur sur les économies ultramarines, en particulier à Saint-Martin, qui dépend très fortement du Alors qu'un nouveau confinement a frappé l'Hexagone, les chances d'une reprise de l'économie saint-martinoise semblent minces. Si notre territoire est épargné par ce nouveau confinement, il en subit de plein fouet les conséquences économiques. Or, trois ans après notre épisode climatique, notre collectivité est toujours en reconstruction et demeure l'une des plus pauvres de France en termes de PIB par habitant.

Aussi, une prolongation des dispositifs exceptionnels d'aide, au moins jusqu'au premier semestre de 2021, sera indispensable pour soutenir notre fragile tissu entrepreneurial.

dont les États-Unis, à la condition d'avoir signé une convention avec l'ARS et la préfecture, engageant ainsi leurs responsabilités. Toutefois, nos attentes en matière de rénovation et de réhabilitation hôtelières demeurent très importantes.

J'espère que l'Assemblée nationale suivra la sagesse sénatoriale lors de la commission mixte paritaire. Monsieur le ministre, vous envisagez de décliner le plan de relance par territoire, en concertation avec les acteurs locaux, ce que je ne puis qu'approuver. Je me réjouis de l'intégration de nouvelles générations ; je pense notamment à la création de la plateforme « Un jeune, une solution ». Les mesures annoncées sont les bienvenues, mais elles nécessiteront un suivi attentif pour être à la hauteur des espoirs suscités auprès de nos concitoyens. Face à un taux de chômage des jeunes très élevé sur notre territoire, et qui risque malheureusement de s'aggraver encore, nous devons intégrer davantage notre jeunesse dans le développement d'entreprises et de filières économiques porteuses d'avenir.

Sur ce point en particulier, comme sur celui de l'hôtellerie, nous avons besoin de votre soutien, monsieur le ministre. Je suis convaincue que l'expérience de terrain et les contacts avec le monde professionnel, associés à une formation adaptée, permettraient à ces jeunes générations de répondre aux besoins d'ingénierie locale ou de création de microentreprises. Enfin, monsieur le ministre, je souhaitais vous demander votre appui pour la tenue rapide d'un « Q4 sanitaire ». Il me paraît absolument indispensable, dans cette période difficile que nous traversons, de nous concerter avec nos voisins de Sint Maarten, notamment pour la mise en place de protocoles sanitaires communs et d'une mutualisation des moyens locaux et étatiques. La parole est à M. le ministre.

un budget dont les crédits augmentent significativement. Permettez-moi, avant de commencer mon intervention, d'avoir un mot de félicitations pour le président Stéphane Artano, qui vient d'être élu ce matin

Leur insularité, leur isolement, leur capacité hospitalière, le climat, la cohabitation avec d'autres épidémies, comme la dengue, ou leurs caractéristiques démographiques sont autant de facteurs qui influent inévitablement sur l'évolution de l'épidémie.

En Guadeloupe, sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l'évolution est favorable, avec des indicateurs qui sont passés sous les seuils d'alerte. À La Réunion et à Mayotte, les indicateurs sont également orientés à la baisse, mais nécessitent une attention En Guyane, nous constatons un effet plateau, avec une incidence qui remonte légèrement. L'État reste particulièrement vigilant en la matière. Nous restons aussi très attentifs à la situation en Polynésie française, qui voit ses indicateurs s'améliorer, mais qui fait face à une dispersion du virus sur ses différentes îles. La réserve sanitaire nationale est fortement mobilisée pour apporter

prochain. Cette rapide description de la situation permet de comprendre à quel point il est nécessaire de continuer à adapter une stratégie sur-mesure, comme nous le faisons pour la pour la Martinique, à l'échelle de chaque territoire, d'associer les professionnels de santé, les élus et l'ensemble des forces vives économiques des territoires concernés aux choix de ces mesures,

consacre à nos différents territoires. Vous le savez, ce budget s'étend sur 31 missions et 94 programmes. Au total, il s'élève à 19,6 milliards d'euros en autorisations d'engagement et à 19,2 milliards d'euros en crédits de paiement. Sur ces 31 missions,

les collectivités d'outre-mer. Ce mouvement s'accélérera l'an prochain, puisque, dans le cadre de la révision de la Dacom, nous vous proposerons de légiférer pour quatre ans. Dès l'an prochain, le volume de péréquation augmentera donc pratiquement de 17 millions d'euros. Pour ce qui concerne la mission « Éducation nationale », les 42 millions d'euros des programmes dédiés à l'enseignement et les 37 millions d'euros du programme « Vie de l'élève » sont particulièrement fléchés vers Mayotte et la Guyane. Il s'agit également d'un engagement du Président de la République. Un rattrapage important s'impose dans ces deux territoires, où l'État assure la maîtrise d'ouvrage de la construction d'établissements scolaires.

le député Olivier Serva. Par ailleurs, le renforcement du dispositif d'investissement productif dans le Pacifique, mieux connu sous l'appellation de neutralisation de l'impôt sur les sociétés pour les collectivités d'outre-mer, a également été adopté, grâce à un amendement des députés du Pacifique ; je pense notamment à Philippe Dunoyer, Maina Sage ou encore Nicole Sanquer.

de limiter à Mayotte et en Guyane la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, afin de tenir compte des contraintes propres à ces territoires dans la gestion des déchets. La coconstruction a, une nouvelle fois, bien fonctionné et nous allons continuer ainsi, notamment au sein de la mission. Concrètement, quel est le contenu de ce budget ? Outre les mesures de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, que M. le rapporteur spécial Georges Patient connaît bien, le Gouvernement a présenté un PLF pour 2021 intégrant la principale partie des 100 milliards d'euros du plan de relance.

Plusieurs chiffres sont à retenir : 50 millions d'euros pour accélérer la construction et la rénovation des réseaux d'eau et d'assainissement. Ce sont des actions essentielles pour nos concitoyens, quoiqu'elles relèvent en grande partie de la responsabilité et des compétences des collectivités locales ; M. Dominique Théophile est revenu longuement sur ce point, et je crois savoir que son appel a été entendu. Nous y reviendrons tout à l'heure au cours de l'examen des 50 millions d'euros sont prévus pour le plan Séisme Antilles, notamment afin de renforcer les bâtiments publics et d'accélérer la mise en oeuvre des programmes en cours. Quelque 80 millions d'euros iront à la transformation de l'agriculture et l'équipement des abattoirs. À ce titre, je me réjouis que, après de longues discussions conduites avec mes collègues Julien Denormandie et Clément Beaune et l'engagement personnel du Président de la République,

Je pense aussi à une mesure que le sénateur Michel Dennemont portera dans le cadre des articles non rattachés. Elle permettra d'augmenter le nombre de logements sociaux et étudiants financés par le prêt locatif social à La Réunion.

Je rappelle à cet égard que la France, fortement contributrice au budget de l'Union européenne, n'est pas pour rien dans la mise en place de ce plan de relance européen. Nous connaissons tous l'action diplomatique et personnelle importante du chef de l'État en la matière.

par des investissements dans le champ des compétences régaliennes, dont certains projets se font attendre depuis bien longtemps, il faut le reconnaître. Je pense au programme immobilier de la justice, aux casernes de gendarmerie et des forces Ainsi, entre les mesures d'urgence économique qui représentent à date 4,5 milliards d'euros pour les outre-mer, le 1,5 milliard d'euros « socle »- et non pas plafond ! -du plan de relance et les crédits React-UE, ce sont

les autorisations d'engagement augmentent de 107 millions d'euros et les crédits de paiement de 93 millions d'euros. Ce programme est très observé en raison de la situation sanitaire, économique et sociale. Nous apportons un soutien aux entreprises par le biais de l'augmentation, à hauteur de

supplémentaires en effectifs qui accompagnent notamment l'ouverture d'une troisième compagnie du régiment du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie, à Bourail. C'est une décision que j'ai prise et à laquelle je tiens particulièrement. Sur le programme 123, « Conditions de vie en outre-mer », les autorisations d'engagement augmentent de 85 millions d'euros, avec trois priorités. La première, je le répète, c'est le logement. Les besoins dans les territoires ultramarins sont énormes. Les particularités propres aux outre-mer-

de la politique du logement. Elle voit ses crédits augmenter de 8,7 %, soit 224 millions d'euros, dont 18 millions d'euros en autorisations d'engagement dédiées spécifiquement aux établissements publics fonciers de Guyane En 2020, les engagements de crédits sur la LBU atteindront la cible programmée, et ce malgré les perturbations liées à la crise sanitaire. C'est le résultat- historique ! -de la mobilisation de l'ensemble des acteurs et d'une stratégie plus claire et mieux territorialisée dans le cadre du nouveau

grande nouveauté de cette mission, directement inspiré d'un rapport rendu par Georges Patient et Jean-René Cazeneuve sur l'accompagnement des collectivités territoriales. Mesdames, messieurs les sénateurs, la décentralisation, la différenciation territoriale et la défense des libertés locales sans s'assurer que la puissance publique locale fonctionne effectivement. Les collectivités ont besoin d'un accompagnement particulier en ingénierie et en matière financière. Les contrats d'accompagnement proposés dans ce rapport sont une réponse pertinente à cet enjeu. Comment fonctionneront-ils ? Nous pourrions commencer, sur la base du volontariat, par identifier une dizaine de collectivités en 2021, avec un objectif : résoudre l'écart structurel entre les recettes et les dépenses. L'idée L'idée est d'avoir des engagements de la collectivité à bien mettre en place des mesures de retour à l'équilibre et d'amélioration de la gestion et de lui proposer, en contrepartie, un accompagnement de l'État et un soutien financier exceptionnel, dont la reconduction sera conditionnée aux résultats.

contractualisation. Enfin, au sein de cette mission, le Gouvernement vous présentera un amendement visant à compléter la réforme engagée de la continuité territoriale. C'est un sujet qui, je le sais, est très important pour les parlementaires ultramarins. C'est d'ailleurs à la suite d'un rapport parlementaire

l'augmentation du montant du bon ACT dans les collectivités d'outre-mer, afin qu'il puisse correspondre à une prise en charge d'environ 40 % du prix du billet, comme dans les DROM, ou encore l'ouverture du passeport pour la mobilité des études à des formations non diplômantes. La majorité des propositions n'est pas de nature législative, sauf celle sur l'élargissement du bénéfice de l'aide obsèques. Un amendement, déposé par le Gouvernement et reprenant la majorité des idées des parlementaires, a pu répondre aux principales attentes exprimées. Cette aide est désormais ouverte aux frères et soeurs des défunts et aux déplacements liés à la fin de vie. Lors de l'examen de la mission à l'Assemblée nationale, nous avons complété l'amendement gouvernemental par une nouvelle proposition parlementaire, preuve que la coconstruction est au coeur de notre méthode de travail. Désormais, l'article 55 , tel tel qu'il vous est présenté, permet d'étendre la mesure de continuité obsèques aux déplacements entre territoires d'outre-mer. Néanmoins, je suis conscient que la disposition est encore perfectible. À la suite d'échanges nourris avec M. le rapporteur spécial Teva Rohfritsch, il est apparu utile de simplifier l'écriture de la mesure, qui, à force de modifications, devenait peu intelligible, et d'opérer deux élargissements supplémentaires, afin de tenir compte de toute la diversité des situations familiales dans les outre-mer. Aussi, l'amendement que M. le rapporteur spécial vous présentera tout à l'heure permet, d'une part, d'étendre la mesure aux trajets des outre-mer vers l'hexagone, d'élargir les conditions d'octroi de l'aide. Ainsi, pour bénéficier de l'aide, le décès ne devra plus avoir lieu avant le voyage aller, comme prévu aujourd'hui, ni avant le voyage retour, comme prévu dans l'article 55 , mais dans les trois mois après le voyage aller. permettra de prendre en compte des situations douloureuses de personnes, qui, parfois, doivent rentrer avant le décès, lequel n'intervient malheureusement que quelques jours après. L'ensemble de ces mesures est estimé, pour 2021, à 3 millions d'euros, qui sont déjà intégrés dans les crédits initiaux de la mission « Outre-mer ». Mesdames, messieurs les sénateurs,

Les mesures contraignantes de quarantaines visant à maintenir tout nouvel arrivant sur le sol calédonien pendant une durée de quinze jours dans des hôtels réquisitionnés à cette fin permettent à ce territoire d'être aujourd'hui « covid protégeant ainsi une population particulièrement vulnérable. Le présent amendement vise à transférer 75,4 millions d'euros de l'action n° 01 vers l'action n° 04, afin de financer par la solidarité nationale les mesures de quarantaine imposées en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui supportées par le seul gouvernement calédonien.

Le soutien de l'État à la politique menée par la Nouvelle-Calédonie repose d'ores et déjà sur un prêt garanti par l'État à hauteur de plus de 28 milliards de francs Pacifique, soit 230 millions d'euros. Par ailleurs, comme pour les autres collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie est éligible au plan de relance. Je sais également que le Gouvernement travaille sur la question spécifique des finances de la Nouvelle-Calédonie, un sujet sur lequel je souhaite entendre M. le ministre.

de vie outre-mer ». La survie des compagnies aériennes des collectivités du Pacifique, qui assurent presque seules la desserte et le désenclavement de ses archipels, est gravement menacée par la crise sanitaire. La compagnie Aircalin représente 80 % du trafic international vers la Nouvelle-Calédonie. Elle joue à ce titre un rôle primordial de continuité territoriale. Pour faire face aux difficultés liées à la crise sanitaire, la compagnie a présenté un plan de sauvegarde et de relance, comprenant notamment une réduction de 20 % de sa masse salariale, et a obtenu un prêt garanti par l'État de 40 millions d'euros. Pour autant, ces mesures sont insuffisantes, et seul un soutien financier spécifique de l'État, comme celui dont ont bénéficié

Je crois l'avoir déjà dit au président Édouard Fritch, je crois l'avoir dit devant vous et je crois l'avoir dit devant toute la délégation qui avait été emmenée devant le Premier ministre et que j'ai reçue à mon ministère.